Madame la ministre,

Je ne dénie pas au Président de la République le droit de laisser l'empreinte de son quinquennat sur la culture par un label